samedi, le matin et l'après-midi uniquement, afin d'aller plus avant dans l'examen des articles non rattachés de la seconde partie du projet de loi de finances. Il n'y a pas d'observation ?

rapporteur spécial des crédits de la mission « Outre-mer » pour la commission des finances. Ne pouvant être présent aujourd'hui, il m'a demandé de le remplacer. Les crédits de la mission « Outre-mer » s'élèvent à 2,5 milliards d'euros en crédits de paiement. C'est l'une des plus petites missions du budget de l'État, mais ses crédits ne retracent que 12 % de l'effort total de l'État en faveur des outre-mer, estimés à 22,05 milliards d'euros en autorisations d'engagement (AE) et à 21,5 milliards d'euros en crédits de paiement portés par 90 programmes relevant de 30 missions. Les dépenses fiscales étant estimées à 4,5 milliards d'euros, l'effort total de l'État devrait s'élever à 26,55 milliards d'euros en AE et à 26 milliards d'euros en CP en 2020. Les principales missions concernées sont la mission « Enseignement scolaire », qui porte 24,8 % de l'effort de l'État en faveur de l'outre-mer,

Hors dépenses de personnels, les missions « Enseignement scolaire » et « Écologie » connaissent les hausses les plus importantes en valeur absolue, tandis que la mission « Outre-mer » connaît la plus forte diminution, soit une baisse de 105,5 millions d'euros entre 2019 et 2020. les crédits alloués à la mission sont en baisse de 1,3 % en AE et de 3,9 % en CP par rapport à 2019. Cette baisse me paraît regrettable dans la mesure où la mission a vocation à favoriser le rattrapage des territoires ultramarins.

Le programme 138, « Emploi outre-mer », rassemble les crédits visant à lutter contre ces forts taux de chômage. Plus spécifiquement, il comporte les crédits visant à compenser aux organismes de sécurité sociale les exonérations spécifiques de cotisations patronales. En 2019, le dispositif d'allégements et d'exonérations de charges patronales dans les outre-mer a été modifié afin de répondre entièrement aux dispositions de l'article 86 de la loi de finances pour 2018, qui a acté la suppression du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au 1 janvier 2019. cette réforme avait entraîné une augmentation de plus de 42 % des crédits affectés à la compensation de ces exonérations de charges. Ces crédits subissent en 2020 une diminution de 2,3 %, mais il semblerait que cette baisse soit purement technique, liée à la fiabilisation en cours des prévisions de compensation par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Sur le fond, je tiens à dire que les nouveaux paramètres du régime issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 n'ont pas permis de pleinement compenser les effets de la suppression du CICE. Au total, la perte nette pour les territoires ultramarins pourrait être de l'ordre de 60 millions d'euros pour l'année 2019, selon les estimations de la Fédération des entreprises d'outre-mer (Fedom).

» et les seuils d'entrée dans ce régime ont été modifiés. De même, dans le secteur aérien, les cotisations de retraite complémentaire seront prises en compte dans le calcul des allégements généraux. Ces mesures permettront de récupérer 35 millions d'euros, même si des progrès restent à faire, s'agissant notamment des entreprises guyanaises. Le programme 138 finance également les crédits du service militaire adapté (SMA), qui constitue un dispositif efficace d'insertion socioprofessionnelle des jeunes ultramarins, puisque 82 % des 6 000 jeunes qui y ont été accueillis se sont retrouvés insérés à l'issue de leur parcours de formation. 2020 verra la mise en place du plan SMA 2025, qui vise à renforcer l'encadrement et à améliorer l'adéquation entre l'offre du SMA et les besoins géographiques, conformément aux préconisations que Nuihau Laurey et moi avions formulées à

L'objectif fixé par le Gouvernement est un taux d'encadrement de 16,3 % en 2022, contre 15,6 % en 2018, mais 22 % en 2010. Dans le domaine du logement, nous indiquons chaque année que les moyens mis en oeuvre restent largement inférieurs aux besoins exprimés par tous les acteurs, publics ou privés. Nous notons pour 2020 une baisse particulièrement importante des crédits alloués, de plus de 3 % en AE et de plus de 13 % en CP. Ces crédits, qui sont malheureusement en baisse chaque année depuis 2014, atteindront en 2020 leur plus bas niveau historique sur les dix dernières années, alors que le déficit de logements est de plus en plus criant dans tous les territoires. En matière de relance de l'activité économique, nous notons avec satisfaction le maintien, en 2020, du fonds exceptionnel d'investissement (FEI) à hauteur de 110 millions d'euros en AE. Je rappelle qu'en 2019 le Gouvernement avait demandé la suppression de 170 millions d'euros de dépenses fiscales en outre-mer. En contrepartie, il s'était engagé à utiliser les gains budgétaires ainsi réalisés pour abonder ce fonds destiné à soutenir le développement économique. Ce choix était justifié par le caractère plus « pilotable » des dépenses budgétaires, qui permettent un meilleur ciblage que la dépense fiscale. Il n'offre cependant aucune garantie quant à leur pérennité. Avant de conclure, je tiens à exprimer ma satisfaction concernant le maintien du prélèvement sur recettes (PSR), qui existe depuis 2017, au profit de la collectivité territoriale de Guyane (CTG). D'un montant de 27 millions d'euros, celui-ci a vocation à compenser les pertes de recettes résultant de la suppression de la part d'octroi de mer de la collectivité. Sa transformation en dotation budgétaire, dont le versement aurait été conditionné au respect d'une convention par la CTG, aurait pu mettre en danger les finances de cette collectivité. Enfin, permettez-moi de relayer la préoccupation de mon collègue Nuihau Laurey s'agissant de la participation de l'État au financement du régime de solidarité de la Polynésie française (RSPF). Cette participation a été supprimée dans l'attente de la mise en oeuvre de nouvelles mesures faisant suite à une mission diligentée par l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) en 2018-2019. Pouvez-vous nous éclairer, madame la ministre, sur l'avenir de ce régime et de son financement ? Au final, la commission des finances, suivant l'avis de ses deux rapporteurs spéciaux, a émis un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission « Outre-mer ». Je vous proposerai donc de la suivre.

Nous avions aussitôt indiqué que les 170 millions d'euros de ponctions fiscales sur les ménages et les entreprises ultramarines pénaliseraient l'activité sur nos marchés économiques étroits. Le Gouvernement s'était alors engagé à reverser le même montant sous forme de subventions. Toutefois, à supposer que cet engagement soit respecté dans le temps, chacun sait ce que cela implique en termes de procédures et de

Or que constate-t-on aujourd'hui ? Les organismes de sécurité sociale anticipent une baisse du recours aux allégements de charge. Cela signifie en clair que l'emploi risque de décliner et que les entreprises ne retrouvent pas dans les nouveaux allégements un dispositif aussi incitatif que le précédent. À cela s'ajoute l'aggravation constante de la sous-consommation des crédits pour le logement, laquelle traduit une diminution de l'effort de construction et de réhabilitation. Loin de progresser vers l'objectif fixé à un niveau raisonnable dans la loi, on s'en éloigne. Attention, les clignotants s'allument s'agissant de la baisse d'efficacité de la dépense publique. On assiste non pas au fameux effet multiplicateur keynésien, mais plutôt à un cercle vicieux : l'insuffisance des recyclages produit des effets récessifs, qui, à leur tour, réduisent la capacité des territoires à activer les crédits budgétaires. Madame la ministre, il fallait absolument réagir tout de suite. J'ai plaidé en commission des affaires économiques pour un rattrapage immédiat dans ce budget des outre-mer. Je rappelle ici que les crédits des outre-mer sont largement déterminés par les mesures adoptées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour paramétrer et le cibler les allégements de cotisations sociales sur certains secteurs économiques offensifs ou exposés.

Nous devons poursuivre ce travail pour rendre les allégements de charges plus performants, car ils jouent un rôle essentiel dans la structuration économique et sociale de nos territoires. On ne peut pas, d'un côté, dire que c'est le manque d'ingénierie qui handicape la construction et, de l'autre, refuser d'en tirer les conséquences et d'aider les entreprises à retenir les talents ultramarins prêts à s'expatrier,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, j'interviens en remplacement de ma collègue Nassimah Dindar, qui me prie de bien vouloir l'excuser. Les crédits de la mission « Outre-mer » ne représentent qu'un peu plus d'un dixième de l'ensemble de l'effort budgétaire assumé par l'État à destination des territoires ultramarins. La commission des affaires sociales est à la fois satisfaite du maintien du niveau des crédits de la mission au-dessus du seuil symbolique de 2,5 milliards d'euros, et réservée sur la lisibilité et la répartition Le programme « Emploi outre-mer », qui concentre plus de la moitié des dépenses de la mission, soit 1,47 milliard d'euros, retrace pour l'essentiel la compensation budgétaire des exonérations de cotisations sociales dites Lodéom, dont bénéficient les entreprises de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion, ainsi que de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Par ailleurs, notre commission, qui a récemment réaffirmé son attachement au principe de la compensation intégrale par le budget de l'État des pertes de recettes pour la sécurité sociale, s'étonne de la baisse du montant affecté à cette compensation. Non seulement cette baisse suscite l'inquiétude légitime des acteurs économiques ultramarins, mais elle ne semble pas tenir compte des mesures incitatives nouvelles inscrites dans le PLFSS. Le programme « Conditions de vie outre-mer » comprend principalement le financement du logement social. Cette ligne budgétaire unique mobilise en 2020 un peu plus de 215 millions d'euros en autorisations d'engagement, soit une baisse de 3,15 % par rapport à 2019. Notre commission a de nouveau alerté avec force sur le niveau et le pilotage des crédits attribués à cet objectif spécifique. Nous serons très attentifs aux orientations données par le ministère, qui entend désormais distinguer les opérations de construction et les opérations de réhabilitation, afin de afin de déployer une politique du logement moins uniforme et plus attentive aux besoins spécifiques de chaque territoire. Néanmoins, nous ne cachons pas notre inquiétude. La situation particulière de la Guyane et de Mayotte, où l'explosion démographique entretient de manière

et social prévus dans le cadre de la présente mission sont disparates et limités, mais ils demeurent des outils essentiels d'appui aux politiques menées par les différents ministères. À ce titre, ils doivent être préservés. Sous ces réserves, et en renouvelant son souhait que les crédits sociaux fassent l'objet d'un pilotage plus fin et plus adéquat, la commission des affaires sociales a émis un avis favorable à l'adoption

En deuxième lieu, le projet de budget ne prend pas en compte le produit de cessions qui viendront abonder la ligne budgétaire unique. Enfin, en troisième lieu, cette baisse s'explique par la sous-exécution récurrente du budget de la mission « Outre-mer Il n'est pas acceptable, alors que nos territoires ultramarins souffrent de retards de développement, que, chaque année, des crédits soient rendus à l'État, faute de projets suffisamment aboutis pour les dépenser. Plusieurs mesures de soutien à l'ingénierie seront mises en place en 2020. J'espère qu'elles seront suffisantes pour que les crédits attribués soient pleinement consommés. La mission « Outre-mer » ne représente par ailleurs qu'environ 10 % des crédits consacrés aux territoires ultramarins. En 2020, ceux-ci sont en augmentation de plus de 15 %. Ces éléments ont conduit la commission des lois à émettre un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission « Outre-mer ». J'ai souhaité aborder plus précisément, à l'occasion de mon avis, l'action du budget de la mission consacrée à l'insertion des collectivités ultramarines dans leur environnement régional. Dans la mesure où cette thématique a fait l'objet de modifications législatives d'ampleur en 2016, il m'a semblé intéressant, trois ans après, d'en faire un bilan. Une bonne insertion de ces territoires dans leur bassin géographique permet en effet aux collectivités à la fois d'affirmer leur potentiel économique, culturel, scientifique et technique, mais aussi de contribuer au rayonnement de la France dans toutes les zones du monde. Le bilan diffère cependant selon les zones et, à l'intérieur de ces zones, suivant les collectivités. De manière générale toutefois, on constate plutôt une sous-utilisation par les collectivités de leurs compétences et des dispositifs de financement existants. Afin d'encourager l'utilisation par les collectivités ultramarines de leurs compétences internationales, une politique de soutien a été mise en place par l'État : ambassadeurs délégués, conférences de coopérations régionales et, récemment, conseillers diplomatiques auprès des préfets

Nous devons également travailler sur l'acceptation des actions de coopération décentralisée par les pays et territoires voisins. Enfin, la coopération décentralisée est pensée pour être réalisée entre collectivités de même taille et aux compétences équivalentes.

local. Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque discussion comprend le temps de l'intervention générale et celui de l'explication de vote. Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de vingt minutes pour intervenir.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les territoires ultramarins souffrent de nombreux maux et les conditions de vie y deviennent de plus en plus difficiles pour nos concitoyennes et concitoyens.

nocifs pour la santé y sont ajoutés, afin qu'elles soient préservées lors de l'importation depuis la France métropolitaine. Ces additifs alimentaires sont particulièrement dangereux et entraînent une surreprésentation des cas d'hypertension artérielle et de diabète dans les territoires ultramarins.

Pour parfaire ce tableau problématique, il faut savoir que les territoires ultramarins ne bénéficient même pas d'infrastructures de soins adaptées pour accueillir les populations particulièrement touchées.

Comment expliquer que, par un amendement déposé à la dernière minute, votre majorité à l'Assemblée nationale ait décidé de raboter encore de 10 millions d'euros ce budget, dont 8 millions d'euros sur le programme « Conditions de vie outre-mer »

Soumis au dogme libéral, l'exécutif estime que le progrès social dans ces territoires passera par une plus grande compétitivité du tissu économique local. Ainsi, le Gouvernement a fait le choix de réduire massivement les cotisations sociales des entreprises ultramarines, au détriment des dotations destinées aux services publics et au logement, Vous l'aurez compris, mes chers collègues, comme les banlieues et les campagnes sur le territoire métropolitain, les outre-mer sont aujourd'hui laissés à l'abandon par les pouvoirs publics. publics. Ne laissons pas les 2,7 millions de Français ultramarins sans aides, avec un pouvoir d'achat très faible. Plus que jamais, ils ont besoin d'un retour de l'État pour redynamiser leur économie et redéployer des services publics là où ils sont inefficients. Les habitants de Mamoudzou, Cayenne et Fort-de-France ont les mêmes droits que ceux de Paris, Lyon ou Strasbourg ! Ils ne sont pas des citoyens de seconde zone. Que le Gouvernement cesse de les traiter comme tels !

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous partageons tous le désir d'aider les outre-mer à relever les défis auxquels ils sont confrontés. Nous avons tous le devoir de parvenir à instaurer une égalité réelle entre tous les territoires, afin que chaque citoyen puisse vivre avec le sentiment d'appartenir à une seule et même communauté. C'est pourquoi le projet de budget pour l'outre-mer revêt, chaque année, un intérêt particulier. Les crédits de la mission « Outre-mer » pour 2020, répartis en deux programmes, consacrés l'un à l'emploi outre-mer, l'autre aux conditions de vie outre-mer, sont en diminution. Ils s'élèvent à 2,56 milliards d'euros en autorisations d'engagement et à 2,41 milliards d'euros en crédits de paiement, soit une réduction de respectivement 3,96 % et 6,45 % par rapport à la loi de finances pour 2019. Cette diminution s'explique en partie par des mesures de périmètre et de transfert. Une fois celles-ci prises en compte, la baisse se limite à 1,30 % en autorisations d'engagement et à 3,88 % en crédits de paiement. Cette diminution est justifiée par le Gouvernement par une adaptation à la sous-exécution récurrente des crédits consacrés aux conditions de vie outre-mer. Alors que le Président de la République a reconnu la nécessité de donner aux outre-mer les moyens de leur développement, il est regrettable de constater que, chaque année, des crédits ne sont pas engagés ... Non : « pas consommés » ! ... Il est important de le souligner, les crédits de la mission « Outre-mer » ne constituent néanmoins qu'un peu plus de 9 % de l'effort financier global de l'État en faveur des outre-mer. Celui-ci s'élève en 2020 à 26,55 milliards d'euros en autorisations d'engagement et à 26 milliards d'euros en crédits de paiement, soit une hausse de respectivement 15,3 % et 17,3 % par rapport à 2019. Cette forte augmentation vient compenser la baisse des crédits de la mission « Outre-mer » et démontre la prise en compte, par le Gouvernement, de la nécessité d'un effort important en faveur des territoires ultramarins. Je voudrais aborder plus spécifiquement l'insertion des collectivités ultramarines dans leur environnement régional et la nécessité de l'encourager. malgré des compétences larges et des politiques de soutien à l'insertion des collectivités ultramarines dans leur environnement régional, ces dernières ne se sont pas encore entièrement saisies des possibilités qui leur sont offertes. Il apparaît ainsi primordial de les inciter à faire usage des compétences dont elles disposent et à recourir aux nombreux instruments de financement existants. Avant de conclure, madame la ministre, je voudrais m'arrêter sur la situation critique du logement. Le logement ultramarin exige des mesures fortes ! Le logement est la base de la vie familiale. C'est aussi un facteur d'attractivité pour les étudiants. Le logement des seniors est également une préoccupation croissante, en particulier aux Antilles, qui connaissent un vieillissement démographique accéléré.

Le budget pour 2020 honore les engagements pris dans le cadre du Livre bleu des outre-mer, qui définit les priorités du quinquennat pour les territoires ultramarins, et des contrats de convergence et de transformation. Il est conforme aux perspectives du plan SMA 2025 et de la Trajectoire outre-mer 5.0. Pour ces raisons, le groupe Les Indépendants votera les crédits de la mission « Outre-mer » du projet de loi de finances pour 2020.

Nous sommes prêts ici à discuter des 2,5 milliards d'euros que porte en affichage cette mission et même à défendre des amendements pour tenter de l'améliorer. Le rituel est bien rodé ; vous nous opposerez sans aucun doute votre ardeur au travail et la pertinence de votre politique, madame la ministre. À mon sens, il est inutile de se lancer dans des débats ésotériques ; je ne parlerai pas de chiffres. Après un temps d'observation, je préfère vous dire le fond de ma pensée sur cette nouvelle politique de l'État outre-mer. Au fond, le débat ne porte pas sur l'existence ou non d'un réflexe outre-mer. Il existe bien : c'est celui de l'égalitarisme forcené. La solidarité nationale se mégote, forçant chacun à trouver son propre salut : en somme, l'individualisme dans toute sa splendeur. Docteure en soupe salée, vous infligez une purge qu'aucun gouvernement n'avait jusqu'alors osé entreprendre.

pas, les marcheurs, tétanisés, spectateurs impuissants des mauvaisetés infligées, ne sont pas entendus lorsqu'ils font remonter l'état des opinions. Ce ministère, bunkerisé dans ses certitudes et droit dans ses bottes, n'arrive donc plus à masquer sa solitude volontaire. Il n'est ni défendu, ni écouté, ni respecté. Chacun peut mesurer que, année après année, sans doute par résignation, le ministère perd tous ses arbitrages et s'isole davantage. Mettez-vous à la place de vos partisans : tous les instruments de politique économique sont, au mieux, rognés, au pire, supprimés.

la circonscription européenne, la Cité des outre-mer. On vide donc des poches qui, vu d'ici, seraient trop pleines. On agite même tous les marronniers des gnomes de Bercy et on fait siennes leurs obsessions en menaçant les acquis sociaux : là, je pense singulièrement aux congés bonifiés ou à la majoration de vie chère. Pour défense, le ministère choisit soit l'attaque, soit la défausse. Ainsi, on attaque lorsque l'on prétend que le financement de notre développement est devenu trop coûteux. Alors, on ligote, on rabote, on coupe, on supprime ... C'est l'autre nom du cartiérisme budgétaire. Plus pernicieuse est en fait la défausse lorsque vous affirmez que l'incapacité subite des collectivités et des acteurs locaux, singulièrement de l'ingénierie locale, est la seule explication aux réductions budgétaires. Cet argument m'est parfaitement insupportable. Jamais donc l'État ne s'interroge sur sa propre responsabilité dans les sous-consommations, notamment le changement de paradigme, passant de la défiscalisation au crédit d'impôt non préfinancé. Je l'affirme : l'État ne s'empresse pas pour accompagner l'avancement des dossiers et les bloque même parfois. Alors, face à la désespérance et à la montée des insatisfactions, on ruse, on enrobe à grands coups de communication. On survalorise la moindre annonce, on lance des « trajectoires », on présente avantageusement des contrats de convergence sous-dotés, on prétend contre l'évidence faire le bonheur des gens par des paillettes et du strass, qui ne sont que de la poudre aux yeux. En cela, je dois vous reconnaître de la cohérence. Vous mettez bien en oeuvre la pierre angulaire de votre politique annoncée en début de quinquennat : la frugalité Ce gouvernement a ainsi annihilé le sens d'une démarche que tous les élus ultramarins portent depuis des décennies. Cette démarche consistait à cranter petit à petit les avancées sociales et économiques obtenues de haute lutte. Au final, j'en arrive à me dire que le ministère se réduit désormais à sa seule capacité à diriger ses préfectures. Quand tout n'est pas recentralisé à Paris, ce sont aux préfets, qui, pour certains, se prennent pour des proconsuls, que revient la tâche de tout régenter. Certains le font même avec zèle et dévouement. Ils « déchoukent » les élus. Ils vont porter la bonne parole en jouant les stars médiatiques. Ils accusent certains d'être incompétents, d'autres d'être de mauvais gestionnaires et les derniers d'être irresponsables. Ils vont dans toutes les réunions publiques, mais décident dans l'entre-soi. Ils n'administrent plus ; ils gouvernent ! Madame la ministre, nous demandons de vraies concertations, une réelle différenciation et une véritable transparence sur la fongibilité des crédits entre collectivités, que vous avez seule engagée. Je suis- il est vrai -amer, mais je suis tout de même prêt à saluer une nouvelle fois votre courage d'avoir assumé la responsabilité pleine et entière de l'État et des autres acteurs privés

Ces mots prennent tout leur sens au moment où nous examinons les crédits de la mission qui regroupe une partie des politiques à destination des territoires ultramarins. Il est en effet difficile de placer dans un même ensemble des territoires situés aux quatre coins du globe, qui ont comme point commun d'être des entités à part entière du territoire national, même si, en dépit de la loi pour l'égalité réelle outre-mer, certains de nos compatriotes persistent à croire que ce sont des entités entièrement à part.

Ensemble, ils représentent environ un dixième du budget global dédié à l'outre-mer, avec 2,5 milliards d'euros en autorisations d'engagement, en diminution de presque 4 % par rapport à l'année dernière, tandis que les crédits de paiement accusent une baisse de 6,5 pour s'établir à 2,4 milliards d'euros. Il faut bien entendu examiner ces chiffres à périmètre constant, puisque certaines mesures concernant la Polynésie française sortent du périmètre de la mission, tandis que d'autres, comme celles qui concernent la Guyane, y entrent. Une fois que ces éléments sont pris en compte, il en ressort que les autorisations d'engagement sont stables, tandis que les crédits de paiement subissent une baisse globale de 4 %, soit 100 millions d'euros. Comment ces chiffres s'articulent-ils au sein des deux programmes ? Tout d'abord, le programme 138, « Emploi outre-mer », qui finance les actions visant à assurer le développement économique et la création d'emplois, connaît une légère baisse due à la diminution des crédits affectés au remboursement aux organismes sociaux des exonérations de cotisations de sécurité sociale Il est en effet important de le rappeler, près de 73 % des crédits de ce programme viennent couvrir la compensation des exonérations Lodéom en faveur des entreprises ultramarines, mais ce dispositif est indispensable pour leur vitalité. L'année dernière, le Gouvernement s'était engagé à compenser la suppression de 170 millions d'euros de dépenses fiscales en outre-mer en orientant les gains budgétaires vers le fonds exceptionnel d'investissement (FEI) et les dépenses visant à favoriser le développement économique des territoires. Le Gouvernement a tenu ses engagements sur ce point, puisque les crédits sont bien fléchés vers le FEI et vers une nouvelle action n° 04, Financement de l'économie. Néanmoins, au sujet des compensations, permettez-moi, madame la ministre, de m'attarder quelques instants sur la situation de mon territoire, de novembre 2017, le Premier ministre s'était engagé à ce que l'État verse entre 2018 et 2020 un appui annuel de 50 millions d'euros par an en fonctionnement, certes assorti de conditions, pour compenser les pertes éventuelles de recettes fiscales faisant suite au passage de l'ouragan Irma. En fait, seuls 25 millions d'euros ont été versés en 2018. Pour 2019, la collectivité vient d'être avisée

À supposer que la collectivité ait pu faire des erreurs de jugement ou de stratégie, cela ne justifie pas pour autant le changement brutal de règles, qui va avoir des conséquences sur la population saint-martinoise et ralentir la reprise de l'activité économique.

Le reste des crédits du programme 138 vient financer le service militaire adapté, qui est particulièrement performant, et l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (Ladom). Ces deux outils en faveur de nos jeunes doivent être pérennisés.

809 millions d'euros en autorisations d'engagement et à 659 millions d'euros en crédits de paiement. L'instrument principal de ce programme est la ligne budgétaire unique (LBU), avec 215 millions d'euros en autorisations d'engagement et 190 millions d'euros en crédits de paiement en 2020, soit une baisse particulièrement forte, de l'ordre de 13 %. Ce niveau constitue le taux historiquement le plus bas de ces dix dernières années. Quand on connaît la situation dégradée du logement en outre-mer, ce choix budgétaire est difficilement compréhensible. Je note enfin que l'action n° 04, Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports, rassemble un montant de 5,6 millions d'euros de crédits, en diminution de 73,6 %. Quelle est la véritable politique que souhaite mener le Gouvernement dans ces matières ? N'avons-nous pas les mêmes droits et le même accès au sport et à culture ?

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, comme chaque année, nous voici réunis pour l'examen des crédits de la mission « Outre-mer ». Comme chaque année, il nous faut répondre à de grandes attentes dans nos territoires, à la hauteur des enjeux auxquels ils font face. Avec 2,5 milliards d'euros en autorisations d'engagement et 2,4 milliards d'euros en crédits de paiement, c'est un budget équilibré qui nous est présenté par le Gouvernement. Il faut le rappeler, le budget total alloué aux outre-mer, à la hausse en 2020, s'élève, tous ministères confondus, à 26,5 milliards d'euros en autorisations d'engagement et à 26 milliards d'euros en crédits de paiement. Dans le détail, la mission « Outre-mer » bénéficie d'un budget résolument tourné vers l'emploi, car elle favorise la formation professionnelle et l'apprentissage et prolonge les engagements en matière de développement économique exonérations de charges sociales, renforcement des zones franches d'activité, aides à la création d'entreprise. Vous le savez, madame la ministre, le Sénat s'est fortement engagé depuis un an aux côtés des socioprofessionnels dans la réforme des exonérations de cotisations sociales. Dans le PLFSS 2020, nous avons, là encore, modifié les paramètres du dispositif. Pour autant, nous devons reconnaître l'effort consenti par le Gouvernement, estimé à 36 millions d'euros, dans la clause de revoyure. De même, chers collègues, reconnaissons, chiffres du chômage à l'appui, l'intérêt d'une telle mesure pour nos territoires et nos entreprises. On ne le dit peut-être pas suffisamment, mais, dans les secteurs renforcés, zéro charge jusqu'à deux SMIC, c'est en définitive 80 % des salaires qui seront entièrement exonérés de charges patronales. Certains souhaiteraient que le dispositif permette le retour au pays de nos jeunes diplômés. Il peut y contribuer. Cependant, ne perdons pas de vue notre priorité commune : lutter contre le chômage. la tendance à la baisse qui se poursuit en 2019, sauf à Mayotte, semble nous dire que nous sommes sur la bonne voie. En Guyane, de 22 % en 2017, le taux de chômage est passé à 19 % un an plus tard.

Je veux insister sur l'une de ses recommandations : lutter contre l'illettrisme. Il s'agit désormais d'une priorité absolue, tant pour les jeunes que pour les adultes ; c'est une condition nécessaire à l'insertion économique et sociale. Nous devons nous y engager pleinement. En cette matière, le SMA joue déjà un rôle fondamental. Aussi, l'on ne peut que se réjouir de voir l'encadrement développé pour améliorer et individualiser le suivi des stagiaires. Ainsi, 127 ETP supplémentaires seront recrutés durant le quinquennat, dont 35 en 2020. Là encore, nous préconisons un renforcement du SMA, au travers d'un meilleur accompagnement des jeunes filles et d'une coopération accrue avec les acteurs de la mobilité. Plus globalement, madame la ministre, j'attire votre attention sur la nécessité d'évaluer les politiques publiques que nous déployons outre-mer, en particulier dans le domaine de l'emploi. La Cnépéom a le mérite d'exister, mais nous savons tous ici que les moyens dont elle dispose restent limités. Ce budget comporte également le programme 123, « Conditions de vie outre-mer

d'un écart de développement particulièrement important entre l'Hexagone et l'outre-mer, sur la base de nombreux indicateurs, comme le PIB par habitant ou l'indice de développement humain. Cette déception n'est d'ailleurs pas étrangère aux mouvements sociaux qui ont secoué certains de nos territoires ces deux dernières années. En Guyane, les manifestants, scandant tous en coeur : « la fusée décolle, mais la Guyane reste au sol ont voulu faire savoir à l'État, mais aussi à toute la France qu'il ne pouvait y avoir sur un même territoire opulence et puissance, d'un côté, sentiment d'abandon et de soumission, de l'autre. Pour ces raisons, un soutien fort et déterminé de l'État est indispensable déterminé de l'État est indispensable aux collectivités territoriales d'outre-mer. Les contrats de convergence et de transformation signés au mois de juillet dernier, dont les crédits augmentent de 5 %, joueront à leur mesure leur rôle. Le FEI, qui est préservé à 110 millions d'euros, y contribue également en restant au service de projets du quotidien un complexe aquatique, un stade, une opération d'assainissement ou d'électrification. Soutenir les territoires, c'est aussi mieux accompagner nos collectivités territoriales. Il faut le dire, en révisant les critères de péréquation, ce budget reconnaît pour la première fois l'iniquité de traitement entre les collectivités locales d'outre-mer et celles de l'Hexagone. Cela se traduira à terme par une augmentation de 85 millions d'euros en faveur des outre-mer d'ici à cinq ans. Dans le prolongement, il conviendra de tirer les enseignements de la mission de nos collègues Georges Patient et Jean-René Cazeneuve sur les finances locales. outre, dans le même esprit, notre groupe sera naturellement favorable à l'amendement de coordination du Gouvernement tendant à rétablir le prélèvement sur recettes relatif à la compensation des recettes d'octroi de mer au profit de la collectivité territoriale de Guyane. Il s'agit là d'une mesure indispensable à la bonne conduite des finances de la collectivité. La question du logement méritera par ailleurs une attention toute particulière. En dépit de besoins criants, les crédits alloués sont malheureusement en baisse chaque année depuis 2014. Si nous convenons tous de leur insuffisance, ils restent fondés sur les capacités d'engagement constatées dans les territoires ces deux dernières années. Cela étant dit, notre priorité est d'inverser la tendance. À cet égard, le rétablissement de l'aide à l'accession à la propriété et à la rénovation de l'habitat est un signal positif. De même, avec 18 millions d'euros supplémentaires en 2020, les crédits des sociétés immobilières d'outre-mer (Sidom) sont au rendez-vous. C'est une bonne chose. Pour rappel, l'État s'est engagé, à l'issue de la conférence du logement outre-mer, à maintenir les autorisations d'engagement de la ligne budgétaire unique au-delà de 200 millions d'euros annuels en 2020, 2021 et 2022. En parallèle, plusieurs actions de soutien à l'ingénierie seront mises en place dès 2020 pour répondre à la sous-consommation des crédits. Une plateforme d'appui aux collectivités devrait d'abord voir le jour en Guyane. Des crédits de la ligne budgétaire unique seront aussi destinés à l'aide au montage de projets. Enfin, l'Agence française de développement (AFD) continuera sa mission d'accompagnement à la maîtrise d'ouvrage à Mayotte et à Saint-Martin. Bien entendu, cela ne suffira pas. En matière de logement, de nombreuses opérations ont pris du retard, trop de retard. Face à ces urgences, il faudra que chacun assume ses responsabilités. Cela concerne, certes, l'État, mais aussi, comme toujours, les élus locaux. les élus locaux. Vous l'aurez compris, notre groupe votera ces crédits, en conscience, et animé de l'exigence que nous fassions toujours plus pour nos territoires et nos concitoyens. La parole

L'examen des crédits de la mission « Outre-mer » est un rendez-vous annuel qui nous permet à nous, parlementaires ultramarins, de nous prononcer sur la concrétisation budgétaire des engagements politiques du Gouvernement dans les outre-mer, à commencer par le Livre bleu des outre-mer et la Trajectoire 5.0. Il permet aussi d'actionner les leviers financiers et fiscaux pour faire face à des problèmes conjoncturels. Nous en avons tous conscience, l'effort de l'État pour les outre-mer ne se réduit pas à cette mission, qui ne représente en réalité que 10 % de l'effort total de l'État. Ce qui m'interpelle dans le budget des outre-mer, ce n'est pas tant le montant total des crédits budgétaires ; ce sont les contours des dispositifs fiscaux, des aides directes et des subventions économiques, sociales, d'équipements que ces crédits permettent de financer. Ces dispositifs sont-ils toujours adaptés aux besoins de chacun de nos territoires ? Fonctionnent-ils ? Pour le service militaire adapté, je réponds « oui je salue le recrutement de 135 personnes en cinq ans, dont 35 en 2020, ainsi que la création d'une nouvelle compagnie à Bourail en Nouvelle-Calédonie. C'est un dispositif essentiel pour l'intégration de nos jeunes en décrochage scolaire et pour notre territoire en général. Je salue également l'augmentation de 10 millions d'euros de la dotation relative au prêt de développement outre-mer, afin de l'étendre aux entreprises situées dans les collectivités du Pacifique. En dépit de ces efforts budgétaires, ce sont les règles de fonctionnement des dispositifs qu'il faut revoir,

Dans un contexte économique fortement dégradé, les aides et les dépenses fiscales pour les entreprises ultramarines sont indispensables. Or, non seulement leur montant a diminué sensiblement, mais les différences de régimes entre les territoires, les doctrines sévères des services fiscaux dans l'interprétation des règles et la longueur des procédures d'agrément découragent les investisseurs.

En effet, il faut plus de deux ans aujourd'hui pour que vos services et ceux de Bercy instruisent un dossier d'investissement défiscalisé dans le Pacifique, contre quelques mois dans les DOM. C'est décourageant, aussi bien pour les acteurs du développement économique que pour les entreprises. Les investisseurs ne vont plus en Calédonie. La défiscalisation est au point mort, même si quelques grosses opérations, comme l'achat en 2017 avions Airbus par Aircalin, permettent d'afficher un niveau élevé de défiscalisation. Les délais de traitement des dossiers par votre administration ne suivent pas.

cela existe dans les DOM, pour ne pas plomber l'intérêt des entreprises métropolitaines à investir dans les entreprises des territoires du Pacifique, fiscalement autonomes. Vous le savez, avec l'incertitude sur l'avenir institutionnel de notre archipel, les investisseurs se font rares. Les banques ne prêtent pas, les acteurs économiques n'investissent pas et mettent leurs économies à l'abri. Alors, si vous ne les encouragez pas, que reste-t-il ? Il y a une vraie réflexion à mener par votre ministère et par Bercy sur ce sujet, afin de rendre claires, lisibles et stables les aides fiscales pour tous les outre-mer. qui est en question, ce n'est pas l'enveloppe budgétaire globale ; ce sont les conditions d'attribution, et notamment les plafonds des revenus, qui ne sont pas adaptés à la vie chère sur certains territoires comme la Calédonie. Cette année, 600 étudiants étaient exclus des bourses sur critères sociaux, donc de la prise en charge à 100 % d'un billet d'avion pour leurs études, alors que leurs familles n'ont qu'un faible reste à vivre. L'incidence budgétaire d'une telle évolution sera minime, mais cela va changer la vie des étudiants. À l'Assemblée nationale, vous avez d'ailleurs assoupli les conditions pour bénéficier de la continuité funéraire et élargi la continuité territoriale à la mobilité au sein d'un d'un même bassin géographique. Cela va dans le bon sens, celui de l'écoute des besoins des Ultramarins. Mais pourquoi ne pas commencer par appliquer la continuité territoriale aux liaisons inter-îles dans les archipels ?

En dehors des contours de dispositifs à améliorer, il y a enfin les zones grises qui demeurent quand on parle des outre-mer, notamment des collectivités à statut particulier. Les collectivités du Pacifique sont exclues à tort de certains dispositifs : des dispositifs fiscaux, mais aussi des fonds, comme le fonds vert ou le fonds de prévention des risques naturels.

Les travaux menés lors de cette conférence ont défini quatre grands axes : mieux connaître les besoins et mieux planifier pour mieux construire ; adapter l'offre aux besoins des territoires ; maîtriser les coûts de construction ou de réhabilitation

La conférence l'a confirmé : l'outre-mer, c'est surtout un besoin de 90 000 logements, ce sont 110 000 logements insalubres, soit 2 % du parc, un parc social vieillissant et 80 % des ménages éligibles au logement social.

la stabilisation de la ligne budgétaire unique (LBU) au-dessus de 200 millions d'euros de 2020 à 2022, d'autre part, la mise en place d'une aide à l'accession sociale et à la sortie de l'insalubrité spécifique à l'outre-mer. À cet égard, la suppression de l'APL accession il y a deux ans fut une erreur que je me réjouis de voir corrigée. J'en arrive à l'examen des crédits de la mission pour 2020. Ils s'établissent à 2,6 milliards d'euros en autorisations d'engagement (AE) et à 2,4 milliards d'euros en crédits de paiement (CP), soit, à périmètre constant, une baisse de 3,9 % en CP et de 1,3 % en AE par rapport à 2019. Les rapporteurs spéciaux de la mission l'ont parfaitement décrit : « Les outre-mer connaissent une situation économique et sociale très défavorable par rapport à la métropole. Le rattrapage de cet écart persistant constitue le défi majeur de la mission " Outre-mer " du budget général de l'État. » À l'examen du budget, force est de constater, madame la ministre, que certains chiffres ne sont pas bons.

niveau le plus bas depuis les dix dernières années. La ligne budgétaire unique est, quant à elle, en baisse de 30 millions d'euros. Le démarrage du plan logement outre-mer 2019-2022 est bien trop timide et l'objectif de construire ou de réhabiliter 10 000 logements par an risque d'être très difficile à atteindre.

Aussi permettez-moi de vous poser deux questions. Cette budgétisation à la baisse ne risque-t-elle pas de porter préjudice aux territoires qui ont vu de très nombreuses entreprises du bâtiment faire faillite ? au mois de décembre 2017, n'explique-t-elle pas en partie cette sous-consommation des crédits ? Nous connaissons tous le parcours incertain d'une demande de financement pour des logements sociaux. De la prise en considération dans les programmes à l'ordre de service autorisant les embuches et les renoncements peuvent être nombreux et les délais inacceptables. Cela s'explique par le fait que chaque dossier est traité en « tuyau d'orgue qu'un comité de pilotage, rassemblant l'État, les maîtres d'ouvrage et les collectivités, valide globalement l'avancée du stock en gestation et reprogramme d'autres opérations pour remplacer celles qui ne peuvent aboutir. La rigidité des règles de procédure n'aide pas. Il faut la simplifier et mettre de l'huile dans les rouages. Madame la ministre, il y a urgence. Je suis d'accord avec vous pour mettre fin à cette sous-consommation des crédits, La création d'un groupe de travail sur ce sujet va dans le bon sens. Les freins doivent être levés dans les meilleurs délais. Notre devoir est de relancer la machine et de redonner confiance aux familles, aux entreprises, aux investisseurs. L'avenir des outre-mer est en jeu.

Madame la ministre, dans une interview accordée à un site d'information, vous avez déclaré : « Ces chiffres n'ont de sens que si nous répondons aux problématiques du quotidien des Ultramarins.

La population ultramarine, celle de La Réunion en particulier, vieillit très rapidement. À Saint-Pierre de La Réunion, la CCAS a dû construire au cours des six dernières années près de 500 blocs sanitaires au domicile de personnes âgées ou handicapées pour un coût total de 3 millions d'euros, main d'oeuvre comprise. Malgré cela, la demande reste forte, et cela n'est pas propre à la capitale du sud. Madame la ministre, les CCAS et le département sont à votre disposition pour étudier les possibilités de financement de ces travaux d'adaptation au vieillissement de notre population.

Madame la ministre, eu égard à la mission de coordination et d'impulsion de votre ministère, il m'importe de souligner que les chiffres de cette mission, largement commentés et interprétés, traduisent en réalité une trajectoire de politique publique qui s'inscrit au-delà de ce seul cadre budgétaire. Permettez-moi donc de m'y attarder dire d'emblée que mon impatience de voir les outre-mer entrer dans le cercle vertueux du développement et sortir de l'ornière du « mal-développement » est toujours aussi grande : elle ne faiblit pas. ne faiblit pas. Nous devons prendre garde à ne pas nous habituer à des difficultés qui, année après année, changent plus de degré que de nature. Année après année en effet, les outre-mer pâtissent des ajustements des gouvernements successifs, générant une instabilité structurelle du cadre économique et fiscal. C'est le cas de la fiscalité de l'emploi, dont les seuils ont déjà été trop souvent révisés et, surtout, recentrés. De fait, regardés isolément, les seuils d'exonération nouvellement nouvellement établis correspondent bien à la répartition salariale des marchés ultramarins. Toutefois, mis en perspective, ils augurent des économies organisées essentiellement autour d'une ressource humaine peu qualifiée. Or le développement suppose de l'encadrement, donc des compétences ; concentrer les allégements sur les bas salaires revient en somme à faire intégralement supporter le coût de la qualification aux entreprises. J'ai déjà eu l'occasion de vous alerter sur les économies d'aujourd'hui qui font les dépenses de demain. Il me semble qu'il est grand temps de mettre en place, non pas seulement un budget, mais une réelle politique publique impliquant tous les acteurs, nationaux et locaux, donnant réellement aux outre-mer les moyens de leur développement. Ce doit être une exigence soutenue, une ambition partagée et une concrétisation déclinée pour chacun des territoires. Bien sûr, on peut noter avec satisfaction les plans de convergences et les investissements en infrastructures qu'ils apporteront dans les collectivités. Ils sont des conditions nécessaires, mais non suffisantes du développement. Peut-être me répondrez-vous par le fameux « réflexe outre-mer » que vous prônez. Permettez-moi de lui préférer la « culture des outre-mer parce qu'il s'agit non pas seulement d'avoir le réflexe, mais plutôt de construire et de nourrir une relation qui s'inscrive dans le long terme. L'État ne devrait avoir besoin de rappel, qu'il soit extérieur ou systématique, pour penser aux outre-mer, ceux-ci devraient faire partie évidente de chacune des politiques publiques, comme ils sont partie intégrante de la République. Scientifiquement, le réflexe est une réaction automatique à un stimulus. L'emploi du terme « réflexe » signe bien l'aveu- au XXI siècle ! -de l'absence d'une culture des outre-mer. Du reste,

prérequis, revendiqué depuis trop longtemps, fût, à tout le moins, dépassé. Il y va du devenir de ces onze territoires et des attentes légitimes de leurs populations. Une réponse à leur incompréhension face aux retards et leur sentiment d'être parfois secondairement considérés doit être apportée. Il est temps ! Je ne peux davantage taire mon impatience alors qu'en 2019 l'État semble seulement prendre conscience des besoins en ingénierie dans les outre-mer, notamment pour l'élaboration des dossiers de financement du logement. Nous en revenons à mon propos précédent sur le financement des emplois qualifiés ... J'aime à citer cet extrait d'une intervention du général de Gaulle en 1960 : « Tandis que le génie du siècle change notre pays, il change aussi les conditions de son action outre-mer. [ ...] Il n'y a pas de politique qui vaille en dehors des réalités ! » Je me réjouis donc, madame la ministre, de vous savoir prête à aller plus loin dans la différenciation territoriale et je partage votre conviction personnelle d'un article unique fusionnant les articles 73 74 de la Constitution. C'était du reste le sens de ma contribution à la journée d'étude « Réforme territoriale et différenciation(s) », organisé ici même en 2015, au cours La différenciation territoriale met en lumière la dialectique de l'unité et de la diversité [ ...] Pour l'outre-mer, la synthèse me semble réalisée par l'article 74 de la Constitution », c'est-à-dire un article unique, socle de statuts à la carte. Sa réécriture devrait permettre de mettre les institutions au service du développement des outre-mer et de faire en sorte que les politiques publiques prennent leur source dans leurs réalités, y compris pour une coconstruction efficace avec l'État. Là encore, à la notion d'adaptation, permettez-moi de préférer celle de pertinence. Après ces considérations d'ordre général, je tiens à saluer de manière appuyée le travail considérable et de très grande qualité de mes collègues Guillaume Arnell, rapporteur coordinateur, Jean-François Rapin et Abdallah Hassani, rapporteurs, sur le second volet du rapport d'information sur les risques naturels majeurs dans les outre-mer conduit par la délégation sénatoriale aux outre-mer que j'ai l'honneur de présider. Ce volet est, comme le précédent, le fruit d'une observation minutieuse de la situation de chacun des territoires et d'une écoute attentive des parties prenantes à la reconstruction et à la résilience de ces territoires. Nous espérons que le projet de loi fera l'objet d'une véritable coconstruction tenant compte de cette approche de terrain. en évoquant Saint-Barthélemy, pour lever une ambiguïté qui a pu naître du projet d'évolution de l'organisation de la gestion et du financement de la sécurité sociale sur notre île. En 2015, il a fallu le passage du Président de la République pour qu'un véritable service de gestion de la sécurité sociale soit mis en oeuvre sur place,

conduisant d'ailleurs la collectivité à abonder le compte soins de ce dernier. À Saint-Barthélemy, la biologie médicale a reculé de trente ans- il faut cinq jours minimum cinq jours minimum pour une glycémie -et la réorganisation des urgences entraîne une limite de capacité au-delà de deux évacuations sanitaires. Voilà deux exemples symboliques de la dégradation de la prise en charge des patients. C'est dans ce contexte que le président de la collectivité a émis le souhait que la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy soit dotée d'une véritable personnalité juridique, d'une part, que, par dérogation, elle se voit confier le versement des dotations aux établissements de santé de l'île, d'autre part. Saint-Barthélemy ne remet donc aucunement en cause son insertion dans le système de solidarité nationale, mais souhaite être impliquée dans un projet de santé local qui tienne précisément compte de sa réalité. Très bien

madame la ministre, mes chers collègues, voilà déjà trois années que j'interviens à la tribune sur le budget de la mission de ladite « Outre-mer J'aurais pu, comme les deux années précédentes, décortiquer ligne après ligne, remarquer, que dis-je souligner, que dis-je dénoncer des lignes budgétaires en baisse sur des sujets regroupés au sein du programme au hautement éloquent et évocateur « Conditions de vie outre-mer ». La logique, avouez-le, voudrait que l'on baisse un budget quand les choses vont mieux.

a été brutalement arrêté, laissant en panne sèche sur le bord de la route plus de 150 familles en Martinique, alors qu'il avait pu en financer 750 en cinq ans.

payer elles-mêmes leur propre sous-développement en lieu et place d'une obligation légitime de solidarité de la République ! J'aurais pu également évoquer le démontage, pièce par pièce, de tout le système de rééquilibrage équitable qui s'appelait TVA non L'an dernier, ces mesures hallucinantes ont démontré, s'il en était encore besoin, le prisme, le regard tronqué, l'angle mort avec lequel on nous regarde, cet angle mort de la République envers ces pays dits « de l'outre-mer ». J'aurais pu poursuivre sur poursuivre sur la baisse manifeste de la LBU, qui acte en budget la politique du logement outre-mer. Oui, les crédits de paiement ont enregistré une baisse. S'est-on posé la question du pourquoi et du comment ? S'est-on posé la question de la souffrance des opérateurs sociaux qui croulent sous les difficultés, certains ayant même préféré mettre la clé sous le paillasson ? J'aurais pu aussi vous dire que nous sommes loin du compte en matière d'exonération de charges sociales, très loin de l'écart creusé, et non rattrapé, par la suppression des mesures énoncées plus haut. haut. Finalement, tout cela est vain. Tout cela et tous les discours n'auraient servi à rien. Un philosophe disait avec justesse que la qualité de la relation que vous entretenez avec un peuple dépend du regard que vous portez sur lui. Eh oui, hélas, c'est de cela qu'il s'agit ! Quand les différents gouvernements, tous, ceux qui vous ont précédé, le vôtre, mais également ceux qui suivront, suivront, considèreront-ils, enfin, que ces territoires ne sont pas simplement destinés à assurer gloire, puissance et splendeur maritime à la France, héritage d'un certain passé ? Quand les différents gouvernements comprendront-ils, enfin, que nous sommes aussi des peuples, assoiffés de jours meilleurs, en quête permanente de conditions d'épanouissement qui riment avec « lutte acharnée contre les dépendances », tendant vers l'autosuffisance aussi bien énergétique qu'alimentaire ? Mais tout cela, avec quels outils ? Avec quel regard ? Avec quelle détermination ? Avec quelle ambition ? voilà pour la troisième fois devant vous, avec l'impression d'être complètement « à côté de la plaque », d'être égarée sur une piste sans issue, dans un labyrinthe inextricable d'impuissance renouvelée et de perception voilée.

héritage fait d'iniquité et d'injustices, héritage de trop d'années d'indifférence, héritage de trop d'années de sous-estimation, héritage de trop d'années de mauvais calibrage, héritage de trop d'années à ne voir en nous que splendeur de l'empire, héritage de variables d'ajustements permanentes et quotidiennes.

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur spécial, madame, messieurs les rapporteurs pour avis, mesdames, messieurs les sénateurs, sénateurs, moi aussi, c'est la troisième fois que je viens devant vous défendre un projet de budget. C'est un exercice important puisqu'il caractérise les grandes orientations du ministère pour 2020.

Ce projet de budget nous donne la capacité de faire encore mieux dans chacun des domaines prioritaires que sont l'emploi, la mobilité, le logement, l'éducation, les infrastructures de base. Je serai amenée à l'expliciter. Le ministère des outre-mer disposera en 2020, à périmètre constant, hors exonérations de charges, de 2,6 milliards d'euros en AE et de 2,5 milliards d'euros en CP. rappelle qu'en 2019 le budget des outre-mer a augmenté de 20 % ; nous maintenons cet effort. C'est un engagement du Président de la République. Je tiens à dire ici, comme je l'ai dit à l'Assemblée nationale

ne veulent pas entendre parler de projets, ils veulent en voir les réalisations- et cela se comprend ! Nous devons, ensemble, être bien plus efficients. Les citoyens nous demandent d'être plus performants : il nous faut l'être ! Oui, les crédits de paiement sont en baisse de 100 millions d'euros- 34 millions d'euros sont liés aux prévisions de l'Acoss sur les exonérations de charges, madame Malet.

en intégrant Mayotte au mode de calcul et en adaptant les critères de répartition pour prendre en compte les charges de centralité de l'enjeu scolaire ainsi que les poches de pauvreté. La solidarité nationale

2020 sera le premier exercice plein de mise en oeuvre des contrats de convergence et de transformation signés avec sept ministres, le Premier ministre et le Président de la République au mois de juillet dernier.

Au-delà de cet appui aux territoires, mes priorités structurantes et celles de mon ministère pour 2020 restent l'emploi et le quotidien des Ultramarins, avec un accent particulier sur la mobilité et le logement.

Nous avons profondément réformé le dispositif d'exonération des cotisations sociales en 2019. Nous sommes allés encore plus loin cette année, en votant la clause de revoyure, comme je m'y étais engagée au Sénat. millions d'euros supplémentaires qui permettront d'exonérer totalement jusqu'à 2 SMIC les salaires des secteurs prioritaires pour nos territoires- tourisme, agrotransformation, innovation

Aujourd'hui, une entreprise qui s'installe outre-mer bénéficie des meilleures conditions pour naître, grandir, investir et embaucher en France. Il ne suffit pas

de cette nature sont aussi à soutenir dans les autres territoires d'outre-mer. L'emploi reste donc le meilleur moyen de changer le quotidien des Ultramarins et d'améliorer leurs conditions Ce n'est pas le seul enjeu, bien sûr, mais c'est une priorité du Gouvernement. C'est aussi la raison d'être du fonds exceptionnel d'investissement, dont les crédits ont été intégralement préservés : 110 millions d'euros

poser la première pierre d'un lycée à Maripasoula, en Guyane, avec vous, monsieur Patient, et d'annoncer la réalisation de la route qui désenclavera cette partie du territoire. J'ai vu et senti à quel point l'État était attendu sur la question des infrastructures du quotidien.

La ligne budgétaire unique n'est au demeurant pas le seul moyen mis à la disposition du logement dans les territoires d'outre-mer. Je rappelle que la défiscalisation dans le secteur du logement social outre-mer représente plus de 230 millions d'euros.

des outre-mer, l'engagement fort d'Action Logement de flécher une enveloppe de 1,5 milliard d'euros dans son plan d'investissement volontaire outre-mer. Action Logement lancera un appel à manifestation d'intérêt dans chaque

Ma priorité, c'est aussi la formation professionnelle en mobilité, pour les demandeurs d'emploi comme pour les jeunes. Nous allons la soutenir vigoureusement. Me permettez-vous, monsieur le président, de répondre très rapidement à plusieurs interrogations

Il s'agit d'un amendement de coordination à la suite de l'adoption, en première partie, de l'amendement n° I-1198, qui rétablit le prélèvement sur recettes (PSR) relatif à la compensation des recettes d'octroi de mer au profit de la collectivité territoriale de Guyane.

Madame la ministre, nous vous offrons une occasion extraordinaire de mettre votre gouvernement au pied du mur et d'inscrire dans le projet de loi de

de septembre 2019, un sans-domicile fixe a été retrouvé mort dans les rues de Fort-de-France, en Martinique. Un mois plus tard, deux sans-abris décédaient à Papara, à Tahiti. Rien que dans les rues de Papeete, 300 personnes vivent dehors, dans une extrême pauvreté, sans toit pour dormir. Ils sont plusieurs milliers à l'échelle de l'outre-mer. Dans de telles conditions, nous pouvions espérer

tant pour construire de nouveaux logements sociaux que pour rénover ceux qui existent déjà et qui sont bien souvent trop insalubres. La situation est passablement catastrophique : le nombre de logements neufs construits outre-mer a baissé en 2019 de 8,6 %. C'est à l'État de donner l'impulsion et d'être à l'initiative de nouveaux projets immobiliers, qui doivent bénéficier aux Ultramarins les plus précaires. Ce n'est évidemment pas en baissant les crédits de l'action n° 01 que nous atteindrons ces objectifs ! Ainsi, cet amendement vise à créer un fonds spécial venant soutenir l'action en faveur du logement outre-mer. Ce fonds serait doté de 10,5 millions d'euros.

La prise en compte des spécificités ultramarines est essentielle à une stratégie de santé publique cohérente dans les outre-mer. Plusieurs facteurs sont à considérer : le contexte climatique tropical, dont découle une prévalence des maladies infectieuses et parasitaires, mais aussi la propagation des épidémies, favorisée par un déficit d'eau potable et un environnement souvent insalubre. (CNCDH), dans son avis sur le droit à la protection de la santé dans ces territoires, a alerté sur la présence d'épidémies telles que la dengue, le chikungunya et le paludisme, notamment à Mayotte et en Guyane. L'impact de ces maladies infectieuses dangereuses devrait être considéré comme une préoccupation majeure parmi les enjeux de santé publique en France. Dans un contexte où la prise en charge médicale de la population ultramarine est largement carencée, les pouvoirs

prélevés sur l'action n° 09, Appui à l'accès aux financements bancaires. Ce fonds devrait permettre d'embaucher du personnel médical spécialisé, de mener des campagnes de sensibilisation et de financer la recherche contre les maladies vectorielles.

Alors que les outre-mer souffrent d'une véritable carence en termes d'investissements et de structures sanitaires, sociales et de loisirs, nous ne pouvons laisser se créer de tels écarts avec la France hexagonale. Les dotations des collectivités et services publics étant en baisse, il nous semble judicieux d'injecter les financements étatiques dans des actions pouvant affecter positivement le quotidien des Ultramarins. Ainsi, le présent amendement tend à créer un fonds de 10 millions d'euros ayant pour but de soutenir l'action n° 04, Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports. Cette mesure serait le fruit d'un redéploiement de crédits initialement accordés à à l'appui à l'accès aux financements bancaires qui ne servent qu'à payer les intérêts des banques. Un tel geste viendrait contrebalancer un budget fortement tourné vers l'investissement, afin de redynamiser économiquement les territoires ultramarins, où le chômage est élevé et l'emploi précaire. Le problème de la pauvreté ne peut être simplement résolu en donnant une activité professionnelle à tous. D'autres paramètres doivent également être pris en compte ; c'est le sens de cet amendement. Un soutien accru à l'action n° 04 du programme 123, « Conditions de vie en outre-mer », pourrait se révéler salutaire pour des territoires dont les habitants souffrent au quotidien de manques sanitaires et sociaux, mais aussi de l'absence d'infrastructures éducatives, sportives et culturelles. Nulle part sur le territoire de la République l'exécutif ne devrait abandonner ses administrés sujets aux inégalités sociales.

participé à l'effort collectif martiniquais qui a permis d'engager un certain nombre d'actions qui montrent déjà des signes encourageants. Mais il faut aussi

Certes, elles bénéficient d'un équivalent du Fonds vert, mais ce n'est qu'une solution transitoire. Comme vous l'avez dit, madame la ministre, nous devons mettre en place un fonds pérenne

Jasmin. Cet amendement a pour objet de prendre en compte les problématiques liées à la biodiversité en outre-mer. Si tout le monde s'accorde sur l'urgence écologique et climatique, il demeure pourtant une absence de coordination des politiques publiques déclinées en outre-mer sur ce sujet. Il s'agit donc, par le fonds d'urgence visé, de décloisonner les initiatives existantes et de définir une politique globale et transversale, spécifique à chaque territoire, en tenant compte de la multiplicité des acteurs publics et privés concernés. L'outre-mer est une réserve pour la biodiversité nationale et mondiale qu'il convient de préserver par une action coordonnée, et le pilotage doit être centralisé directement par le ministère des outre-mer. Deuxième domaine maritime mondial, la France héberge 10 % de la biodiversité de la planète, dont la majeure partie en outre-mer. Par exemple, sur 19 424 espèces endémiques recensées, les quatre cinquièmes se trouvent dans les outre-mer

une priorité gouvernementale. L'action n° 02 du programme 138, « Emploi outre-mer », vise à favoriser l'insertion et la qualification professionnelle des jeunes d'outre-mer, notamment grâce à l'accompagnement du service militaire adapté

? Ces amendements ont des objets différents et présentent tous un intérêt certain pour les territoires concernés.

Le programme « Cadres de Mayotte », les chantiers de développement local pour la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie et le programme « Cadres pour Wallis-et-Futuna » verraient ainsi leurs crédits réduits. De même, les ambitions du plan SMA 2025, qui doit notamment permettre une amélioration du taux d'encadrement, s'en trouveraient très largement compromises. La commission des finances a donc émis un avis défavorable à l'ensemble de ces amendements.

sur l'ensemble du Gouvernement pour que ces crédits soient au rendez-vous de 2020. Je sais que vous serez tous très vigilants sur cette question, mais je vous demande de me faire confiance. Vous l'avez compris, nous